par laquelle elle se démet de son mandat de sénatrice du Nord, à compter du lundi 3 juillet. Quel dommage ! Je voudrais saluer la manière dont Mme Blandin a accompli son mandat de sénatrice

En application de l'article L.O. 320 du code électoral, elle est remplacée par Mme Anne-Lise Dufour-Tonini, dont le mandat de sénatrice du Nord a commencé le mardi 4 juillet 2017, à zéro heure. Au nom du Sénat tout entier, je lui souhaite la plus cordiale bienvenue.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, hier, M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur vous a, comme le veut la coutume, donné lecture de ma déclaration de politique générale. Au lendemain du vote de la confiance par l'Assemblée nationale, je ne pouvais qu'être devant vous aujourd'hui, dans cet hémicycle, pour m'adresser directement à vous. N'ayant pas eu le privilège de siéger parmi vous, je n'ai pas le plaisir de tous vous connaître. Sans doute ... Certes, des visages sur ces travées me sont familiers et même amicaux. Certains ont jalonné mon parcours, d'autres m'ont aidé à le construire. Et je ne parle pas seulement de ces grandes figures de notre histoire politique- Victor Schoelcher, Victor Hugo, Georges Clemenceau ou, permettez-moi de le citer, le Havrais René Coty -dont les voix et les intelligences ont fait vibrer ces murs. J'ai par ailleurs l'honneur de compter dans mon gouvernement d'anciens membres de votre assemblée. Les meilleurs ! Le Sénat se confond avec la République. Il en est un pôle d'équilibre. Il est à la fois en prise directe avec le quotidien de millions de Français et à l'écart d'une certaine fébrilité politique. Cette sérénité démocratique est une chance. Hier, dans mon discours, j'ai commencé par rendre hommage à de nouveaux députés qui, par leur parcours, ont remodelé le visage d'une partie de la représentation nationale. Je sais que, comme vous, ils auront à coeur de nouer un dialogue fructueux pour faire avancer le travail parlementaire et pour faire réussir la France. Si je les mentionne de nouveau aujourd'hui, c'est que je m'adresse à une assemblée qui, durant vingt et un ans, a confié sa destinée au petit-fils d'un esclave. Elle l'a fait à une époque où les préjugés étaient encore plus rudes et encore plus injustes que de nos jours. Vos prédécesseurs n'ont pas choisi Gaston Monnerville pour ses origines, mais pour ses talents, ses talents, lesquels n'auraient pu s'épanouir si la République ne les avait pas reconnus et encouragés. C'est de cette République, de cette France de l'égalité des chances, que je veux vous parler aujourd'hui, une France qui, dans les moments les plus difficiles de son histoire, a toujours été capable d'étonnants sursauts. Cette France s'est exprimée durant la campagne présidentielle. Elle a exprimé sa colère, mais elle a aussi exprimé son optimisme et sa volonté de rassemblement. Avant-hier, devant le Parlement réuni en Congrès, le Président de la République nous a montré le cap : celui-ci est clair et sera tenu ! Les Français ont d'ailleurs, dans un souci de cohérence, donné au Président et au Gouvernement une majorité claire et incontestable au sein de l'Assemblée nationale.

Parmi ces devoirs figure évidemment la nécessité de respecter les institutions démocratiques. J'y veillerai. Mais la France doit avancer. Dans « notre cher et vieux pays », il existe une envie, une énergie, un espoir qui transcendent les courants politiques. Le Gouvernement veut s'appuyer sur cette envie et cette énergie pour que la France retrouve confiance : j'ai eu l'occasion de le décliner hier, confiance en son action publique, confiance en sa justice, en sa sécurité sociale et en sa cohésion territoriale. Je veux m'appuyer sur cette énergie pour que, collectivement, nous fassions preuve de courage : courage devant les menaces terroristes et tout ce qui peut menacer la sécurité des Français ; courage devant le défi migratoire pour être fidèles à nos idéaux comme à nos responsabilités pour préparer l'avenir de nos enfants en refondant l'école, pour rénover notre modèle social- il en a besoin -, pour réduire la dette et la dépense publique- c'est indispensable. Je veux m'appuyer sur cette énergie pour que la France redevienne conquérante, pour qu'elle redevienne une terre d'accueil des compétences, des entreprises, des investissements et des intelligences, pour qu'elle restaure la puissance de son agriculture, qu'elle saisisse la chance de la transition écologique et qu'elle assume pleinement sa vocation européenne et internationale. Hier, j'ai indiqué la feuille de route du Gouvernement, son calendrier, sa méthode. Je les résumerai en quelques mots-clefs : la collégialité, la sincérité, la recherche permanente de l'efficacité, et non de la popularité.

il n'est pas impossible que, durant trop longtemps, notre pays ait pris la mauvaise habitude de s'arranger un peu avec la vérité. La Cour des comptes, avec ses mots, nous en a donné une triste illustration. J'y vois une des causes de la crise de confiance qui a secoué notre pays. La vérité n'est pas bâtie dans l'antre des ministères et au sein des cabinets ministériels. Elle se construit et se constate parfois

sur ceux des sujets qui structurent l'avenir du pays. C'est le sens des États généraux de l'alimentation et de l'agriculture, des assises de l'outre-mer, des États généraux des comptes de la Nation et, j'y reviendrai, de la Conférence nationale des territoires.

Je veux donc associer des phases de discussion à l'extérieur des assemblées à d'intenses phases de délibération à l'intérieur de celles-ci. Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne veux pas vous infliger une seconde lecture de ma déclaration de politique générale Ce serait malvenu ! Je ne veux pas non plus vous en infliger une lecture abrégée et commentée, vous n'en avez pas besoin. Non, je veux profiter de ma présence ici pour aborder deux sujets qui vous tiennent à coeur, deux sujets sur lesquels j'ai des choses à dire et, j'en suis sûr, des choses à apprendre de vous. Le premier sujet est institutionnel. Je crois au bicamérisme. Je mesure le rôle du Sénat dans le bon fonctionnement de notre démocratie, et c'est un ancien député qui vous le dit

Mesdames, messieurs les sénateurs, j'y ai toujours cru, mais j'y crois plus encore aujourd'hui, ... - ce qui est en effet déjà considérable ... mais parce que le bicamérisme prend plus encore son sens aujourd'hui qu'hier. D'un côté, nous avons une Assemblée nationale profondément renouvelée. Ce renouvellement était nécessaire. Il était voulu par les Français. Il a été démocratique, clair. Il est une chance pour notre pays. De l'autre côté, nous avons un Sénat où siègent « des élus élus par des élus des élus qui connaissent mieux que personne la réalité des territoires de la République et qui incarnent une expérience des territoires et du processus législatif. renoncé depuis longtemps aux clivages artificiels. On y pratique le sens du consensus et du compromis. On y aime la discussion, le dialogue. On sait y marier les bonnes volontés. Le Sénat, de ce point de vue, a probablement largement anticipé la logique que nous connaissons aujourd'hui. Cette expérience, nous en aurons besoin pour préparer les réformes constitutionnelles dont le Président de la République a dessiné les contours avant-hier, devant le Parlement réuni en Congrès. Réduction d'un tiers du nombre de parlementaires, limitation à trois du nombre de mandats successifs, suppression de la Cour de justice de la République, refonte du Conseil économique, social et environnemental, évolution du travail parlementaire pour le rendre plus efficace et, quand cela est nécessaire, plus rapide : ces réformes seront d'une ampleur dont je ne sais si elle est inédite, mais qui, à l'évidence, sera considérable. Le Sénat, sous l'impulsion de son président Gérard Larcher, a pris les devants. Le 11 mars 2015, votre conférence des présidents a adopté 46 mesures qui ont conduit à une modification du règlement du Sénat le 13 mai 2015 et qui ont en particulier valorisé le travail en commission. Cette expérience, vous aurez l'occasion de la faire valoir par l'intermédiaire de votre président dans le cadre de la réflexion qui s'engage avec le président de l'Assemblée nationale, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, et la garde des sceaux. J'y serai pour ma part très attentif.

mais aussi des usages et des règles qu'adoptent les assemblées et qui fonctionnent bien. Le second sujet que je voulais aborder avec vous concerne l'organisation territoriale de notre pays.

prêtes. Nous voulons que les collectivités locales soient fortes et libres : libres de s'organiser en développant des communes nouvelles ou des regroupements de départements à condition, bien sûr, que ces fusions ne soient pas contraires à l'intérêt général libres d'exercer de nouvelles compétences ; libres aussi de mieux se les répartir au moyen, par exemple, du mandat de délégation libres d'expérimenter non seulement de nouvelles organisations et de nouvelles compétences, mais aussi de nouvelles règles d'exercice de ces compétences dans le cadre d'un élargissement du pouvoir réglementaire local. Liberté et confiance, tels sont les deux fondements de la décentralisation d'aujourd'hui. Une décentralisation qui ne se décrète plus depuis Paris, mais qui s'expérimente, se teste et s'adapte.

pour tendre partout où cela sera possible vers deux niveaux d'administration locale en dessous du niveau régional. Ce ne sera pas le même schéma partout. Essayons de susciter parmi les collectivités, leurs élus, les discussions qui nous permettraient, le cas échéant, à tel endroit de privilégier tel ou tel interlocuteur, à tel endroit, et librement, de privilégier telle ou telle autre organisation. Cette simplification répond à une exigence de bonne gestion. Elle répond aussi à une exigence de lisibilité : l'empilement actuel n'est pas toujours compris de nos concitoyens. Bien évidemment, cette liberté s'accompagnera de solidarité. Une solidarité qui s'exprime d'abord, au niveau de l'État, au travers de la création d'un ministère de la cohésion des territoires dont le titulaire est issu de vos rangs. Cette solidarité s'exprimera aussi par de grands chantiers sectoriels. Dans le domaine de la santé : j'ai demandé à la ministre de préparer pour le mois de septembre un plan de lutte contre les déserts médicaux. Je sais que le Sénat a beaucoup travaillé sur ce sujet crucial sur ce sujet crucial pour l'égalité entre nos territoires. Ce plan sera construit dans le dialogue avec les élus locaux et les professionnels de santé pour trouver des solutions adaptées à chacun des territoires.

et de meilleures relations avec ceux qui défendent les intérêts des professions médicales, nous pouvons cependant faire en sorte d'améliorer cette répartition et de créer des mécanismes incitatifs pour que, au fur et à mesure de notre action, la question,

Dans le domaine de la mobilité : dès la rentrée, se tiendront également des assises de la mobilité. Elles associeront les usagers, les opérateurs, les collectivités territoriales et les associations engagées

élaborer une programmation financière soutenable qui fera porter l'effort non plus sur les grandes infrastructures, mais sur l'entretien et la rénovation des réseaux actuels, la rénovation des réseaux actuels, qui, de toute évidence, ne sont pas satisfaisants. Autre chantier sectoriel sur lequel le Sénat est devenu un expert : le numérique. Comme je m'y suis engagé hier, je souhaite un accès garanti pour tous et partout en France au très haut débit au plus tard en 2022. Mais, là encore, gardons-nous de raisonner uniquement en termes d'infrastructures. Pensons service service à l'usager, service aux collectivités. Cette politique d'accès au numérique nous permettra de déployer de nouveaux projets : je pense notamment au « compte citoyen en ligne » qui pourrait devenir l'interface de base, la norme, entre les administrations et le citoyen. dernier chantier concerne la revitalisation des petites villes et des bourgs-centres, trop longtemps négligée par les politiques publiques, alors qu'elle mérite à la fois une attention particulière et une stratégie propre à chaque territoire : la situation n'est pas la même en Alsace que dans le Massif central, ou en outre-mer. Ces chantiers tendent vers un objectif : combler le fossé qui se creuse entre deux France que certains voudraient opposer, entre deux France qui se vivent parfois comme étant en opposition,

C'est tout l'objet de la Conférence nationale des territoires que le Président de la République a souhaité constituer et dont la première réunion se tiendra mi-juillet. Si vous en êtes d'accord, celle-ci pourrait justement se tenir au Sénat. Ah ! M. le président du Sénat pourrait y tenir le rôle éminent qui lui revient. vous serez évidemment représentés de façon permanente au sein de cette instance par ceux que votre assemblée aura désignés. Un dernier mot peut-être sur les aspects financiers. Je l'ai dit hier, la situation de nos finances publiques est plus que préoccupante, elle est grave. Nous devrons tous contribuer à l'effort de redressement. Je sais que les collectivités locales y ont déjà contribué,

Je crois à la responsabilité des élus locaux, comme je crois à leur sens des réalités. Ils gèrent des budgets, parfois dans des conditions difficiles. Ils sont amenés à faire des choix, à assumer et parfois à revoir leurs priorités. Je sais aussi que « faire avec moins » peut parfois- pas toujours ! -conduire à « faire mieux », c'est-à-dire à proposer des services plus simples, plus agiles et plus efficaces. Nous ouvrirons le dialogue avec les élus pour bâtir une trajectoire commune de maîtrise de la dépense publique. Nous engagerons également la réforme de la taxe d'habitation d'ici à la fin du quinquennat.

des propos que j'ai tenus hier. Je sais cette réforme attendue par les contribuables, mais redoutée par les élus. Alors, parlons-en. Parlons-en avec le Sénat et avec le Comité des finances locales pour réformer cet impôt, qui n'est pas le plus juste, sans porter atteinte à l'autonomie financière des collectivités territoriales. Ce sujet fiscal comme celui de la dépense publique seront évidemment au coeur de la prochaine Conférence nationale des territoires. Au-delà de la taxe d'habitation, je crois pouvoir dire ici que les élus locaux, que les sénateurs encore plus que les élus locaux ont parfaitement conscience du caractère globalement insatisfaisant de la fiscalité locale.

du crâne d'un spécialiste, que je ne prétends pas être. Mais là encore, dans nos échanges, dans nos travaux collectifs, nous pouvons partager ce constat et peut-être lancer ces réflexions au long cours

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je connais comme vous les limites du politique, mais je ne crois pas à son impuissance. Je sais ce que peut la

nous sommes tous frappés par le contraste saisissant qui existe entre le constat souvent dressé d'un pays qui serait bloqué, comme arrêté, et l'incroyable transformation d'un certain nombre de nos territoires

Ils ont choisi de s'attaquer au chômage et de maintenir les fondamentaux de notre République sociale. Ils ont approuvé une stratégie de dédramatisation et de fertilisation de la vie politique, en répondant au président Macron qu'il fallait effectivement dépasser les anciens clivages entre droite et gauche pour plus d'efficacité. Les Français nous invitent à privilégier ce qui nous rassemble et nous commandent d'obtenir des résultats.

Nous devons tout autant reconnaître l'absolue honnêteté et le formidable travail de nos élus sur tout le territoire. Faire progresser la transparence, oui ; l'inquisition, non

Nous soutiendrons la loi quinquennale de programmation des moyens de la justice, la création de 15 000 places supplémentaires de prison et la réforme constitutionnelle renforçant l'indépendance des magistrats.

Nous avons envie de vous soutenir sur ces sujets, mais la promesse d'une réduction de la fracture territoriale et d'une lutte contre les déserts médicaux nous a souvent été faite ...

de répondre à cette attente colossale d'une très grande partie de la France, de remédier à un sentiment politiquement destructeur puisqu'il renvoie vers les extrêmes. thématique est celle du courage. Nous sommes favorables à la sortie de l'état d'urgence au 1 novembre, à condition, bien sûr, de muscler l'arsenal législatif contre le terrorisme et l'insécurité, et de simplifier les procédures administratives imposées aux forces de sécurité.

vous, nos constats sur l'école et l'enseignement sont parfois négatifs : absence de maîtrise de l'écriture et de la lecture, instabilité des organisations scolaires, baccalauréat désuet, échec important à l'université. Les solutions que vous avancez, monsieur le Premier ministre, sont intéressantes. Nous vous suggérons d'aller plus loin, de frapper plus fort, plus définitivement, et comme pour la santé, d'envisager un véritable parcours de réussite scolaire pour tous, qui pourrait aussi commencer par une loi sur l'éducation parentale. Nous approuvons également l'idée d'un nouveau service national pour tous. Sur le modèle social, monsieur le Premier ministre, vous auriez pu choisir de commencer par la phrase suivante : « Les Français souffrent », ceux qui n'ont pas d'emploi comme ceux qui ont un emploi peu ou mal rémunéré. La rénovation sociale que vous proposez en quatre points- dialogue social, pouvoir d'achat, sécurisation des parcours professionnels, système de retraite plus juste -est pertinente. Concertez et, là aussi, essayons d'aller vite ! Un point essentiel, il n'y a pas d'autre voie, et c'est ce que vous proposez, que de rendre du pouvoir d'achat aux Français. Sans

sans efficacité réelle sur l'emploi, la redéfinition du périmètre des politiques publiques et, surtout, la réduction drastique du nombre- surréaliste -d'agences de tout poil et de comités Théodule existant dans notre pays.

pour l'accélération des procédures. Mais vous devriez prendre l'engagement de diviser par deux tous les délais administratifs conditionnant des réalisations dans ce pays : permis, recours, autorisations, enquêtes, etc. Notre pays va à un train de

sommes aussi farouchement déterminés à ce que notre pays se montre plus ferme envers nos amis et partenaires allemands, et tout aussi ferme dans la négociation du Brexit avec nos amis et alliés britanniques.

personnalités de gauche très connues comme Robert Hue et Pierre-Yves Collombat. Ce groupe étant pluraliste, une minorité de nos membres ne partage pas la position que je viens d'exprimer.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues,

Aussi, le groupe Union Centriste ne souhaite qu'une chose : le succès du Gouvernement et la réussite de la France. Nous le souhaitons d'autant plus le projet porté par le Président de la République et le Gouvernement est globalement conforme aux valeurs centristes. Pour que ce quinquennat réussisse, des réformes structurelles s'imposent, celles-là mêmes qui, trop souvent, ont été ajournées, différées, diluées. Force est de le reconnaître : ces réformes sont à l'agenda du Gouvernement, selon des modalités qui suscitent, certes, des interrogations ou qui appelleront de notre part des propositions. Mais, dans ses grandes lignes, monsieur le Premier ministre, nous souscrivons au programme présenté. Dans les quelques minutes qui me sont imparties, il m'est impossible d'embrasser un champ aussi large que celui que vous Nous aimerions aussi pouvoir parler de santé, de retraite, de handicap, de numérique, d'outre-mer, de culture, de sécurité ou d'innovation, sujets sur lesquels nous nous rejoignons très souvent. Je me concentrerai donc sur les réformes qui, à nos yeux, sont les « réformes socles ». Ces mesures sont de deux ordres. Les premières parent au plus urgent. En effet, l'état d'urgence n'est pas seulement sécuritaire ; il est aussi économique et social : nous devons relancer la croissance et l'emploi. La France ne peut rester plus longtemps à la traîne d'une reprise qui s'est intensifiée partout ailleurs. Pour répondre à ce défi, nous pensons comme vous, monsieur le Premier ministre, qu'il faut alléger les charges pesant sur la production et flexibiliser les conditions d'emploi.

Voilà le type d'interrogations que nous avons aujourd'hui et que nous soulèverons lors du débat à venir, dans quelques jours. En contrepartie de la flexibilisation du droit du travail, nous devons garantir des droits aux salariés tout au long de leur vie professionnelle, en particulier en matière de formation. Mais là encore, une question se pose : peut-on réformer la formation professionnelle sans traiter du problème de fond, tabou s'il en est, du financement du syndicalisme salarial et patronal ? Absolument La relance de notre économie est également conditionnée par la maîtrise de nos comptes publics. Le rapport de la Cour des comptes, comme vous-même, monsieur le Premier ministre, vient encore de rappeler que nous n'en avions pas fini avec les déficits

Il n'y aura pas de retour de la croissance et de l'emploi, pas de rétablissement des marges de manoeuvre de l'État, ni d'efficacité de la dépense publique sans assainissement des comptes publics. La technique du rabot a montré ses limites depuis plusieurs années. C'est la raison pour laquelle notre groupe vous accompagnera dans les efforts courageux, notamment de maîtrise de la masse salariale de la fonction publique, que vous avez annoncés.

nous sommes fondamentalement européens. Nous sommes pour une Europe plus forte, mieux intégrée, une Europe qui protège, et ce même si le dernier Conseil européen a démontré à quel point la tâche était ardue en la matière. Nous avons aussi besoin d'une Europe à l'offensive pour défendre

des territoires, nous ne pouvons que soutenir les lignes de force de votre action : expérimentation, liberté, réduction du millefeuille, délégations entre collectivités, couverture numérique, lutte contre les déserts médicaux.

Nous ne demandons pas seulement des compensations ; nous demandons plutôt des recettes dynamiques et pérennes. C'est cela qui permettra d'assurer l'autonomie, que vous avez rappelée voilà quelques instants, des collectivités locales. Vous l'aurez compris, monsieur le Premier ministre, sous réserve de ces interrogations, des propositions que nous formulerons et du traitement qui leur sera réservé, nous abordons ce quinquennat avec confiance, et avec la conviction d'un quinquennat enfin utile.

Je veux donc dire très clairement, au nom de mon groupe, que le tiers payant est une belle mesure de justice sociale et d'équité républicaine,

cause. S'agissant du fond de la réforme du code du travail, vous avez évoqué la sécurisation des parcours professionnels. Il s'agit pour nous d'un point essentiel de la prochaine réforme. Il ne peut y avoir d'assouplissement de certaines règles sans contrepartie forte en termes de protection des travailleurs. La précédente majorité avait créé le compte personnel d'activité. Ce n'est qu'une étape ! Il faut continuer

Nous saluons l'augmentation annoncée de la prime d'activité, le coup de pouce aux salaires et la suppression des cotisations sociales. Mais permettez-nous une remarque : nous pourrons certes soutenir- sans réserve, en ce qui me concerne -l'augmentation de la CSG en parallèle de la baisse des charges, nous nous opposerons à cette augmentation pour les retraités et les personnes âgées. Il n'est pas possible que les retraités moyens soient taxés dans ce cadre-là. Il faut impérativement pouvoir y revenir. Vous avez précisé à l'instant le calendrier de la suppression de la taxe d'habitation. C'est l'impôt le plus injuste. Cela fait un demi-siècle que les bases n'ont pas été revalorisées, personne n'ayant eu le courage de le faire. Elles ne le seront donc jamais. Aussi, la suppression de la taxe d'habitation pour 80 % de nos concitoyens est une bonne réforme. Pas pour les collectivités locales ! Il faut évidemment penser aux contreparties pour les collectivités locales, mais je pense aussi aux 36 millions de Français qui gagneront en pouvoir d'achat grâce à cette mesure. Notre

Monsieur le Premier ministre, vous souhaitez faire des économies : nous vous soutiendrons. Baisser la dépense publique, oui ! Mais maintenir les services publics, trois fois oui ! On ne peut pas réduire les budgets de fonctionnement et réduire les services publics.

comment rapprocher l'Europe des peuples ? Comment faire que les peuples retrouvent confiance dans l'Europe ? Sans doute en donnant un projet politique ambitieux aux institutions. C'est un enjeu majeur, que notre groupe veut accompagner. Lundi, à Versailles, comme à chaque occasion depuis son élection, le Président de la République a prononcé un plaidoyer dans ce sens. dans ce sens. Il faut le soutenir, il faut aller plus loin, sur les questions de défense, sur la protection sociale, sur les travailleurs détachés, sur la zone euro. La liste est longue. Démontrons à nos concitoyens que l'idéal européen est toujours notre horizon.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les membres du Gouvernement, mes chers collègues, lundi dernier, devant le Congrès, le Président de la République a dit une chose assez juste : « Il y a en chacun de nous une part de cynisme, contre laquelle il faut lutter. » Disant cela, il appelait les parlementaires à agir, sans arrière-pensée, dans le seul intérêt du pays. Alors chiche, monsieur le Premier ministre ! Mais pour cela, il y a des préalables. Le premier, c'est le respect de l'opposition. Ni à gauche ni à droite nous ne sommes les deux bouts de l'omelette qu'il s'agirait de réduire pour ne conserver que la partie centrale, fût-elle importante aujourd'hui. Contrairement à certains, je ne vois ici, sur toutes les travées, que des représentants de la Nation. Il n'y a pas d'un côté des constructifs, ... Ah ! ... de l'autre des démolisseurs ; il n'y a ici que des parlementaires disposant du droit et du devoir de contrôler l'action du Gouvernement, du droit d'amendement des textes, du droit de proposer des lois. Ces droits, nous entendons les exercer pleinement. Très bien ! Le second préalable, c'est le respect des Français et de la parole donnée.

D'ailleurs, je suggère qu'à l'avenir nous demandions à la Cour des comptes un audit six mois avant les élections, et non pas juste après pour justifier, à peine élu, l'abandon du calendrier des promesses électorales. Pourtant, le candidat Emmanuel Macron était l'un de ceux qui pouvaient le moins ignorer cette situation, pour avoir été, pendant quatre années, au coeur du pouvoir. Certes, il a plaidé pour le rétablissement de nos comptes publics et l'inversion de la courbe de la dette, qui va finir par nous entraîner par le fond. Certes, il a posé le problème de la compétitivité de nos entreprises et annoncé une hausse de la CSG-ce n'était pas notre choix -pour financer des baisses de charges, pour les entreprises comme pour les salariés, et la fin du CICE dès 2018. Certes,

les Français ont eu droit à une liste de promesses toutes plus sympathiques les unes que les autres, jusqu'à, cerise sur le gâteau, la suppression de la taxe d'habitation pour 80 % d'entre eux, ce qui coûtera 10 milliards d'euros par an. Sur l'équilibre de notre système de retraite, aucun besoin, disait Emmanuel Macron en campagne, de toucher à l'âge de départ à la retraite. On unifierait les différents régimes sans toucher au montant des pensions, et les conséquences de tout cela seraient reportées au-delà de cinq ans, soit après 2022, ce qui doit être une heureuse coïncidence de calendrier ... Seulement voilà, patatras ! Le Conseil d'orientation des retraites vient de le contredire, réaffirmant que, sans nouvelle réforme, la situation continuerait de se dégrader, ce qui reporte aux calendes grecques le règlement du problème. La semaine dernière, la Cour des comptes a rendu son audit dénonçant un dérapage de 8 milliards à 9 milliards d'euros du budget 2017, rappelant combien la situation de nos comptes publics est dégradée, laissant la France à la remorque de quasiment tous les pays européens. Monsieur le Premier ministre, vous nous avez surpris en feignant de piquer une colère et en vous exclamant : « Comment cela ? On nous avait donc caché des choses ? » Ainsi, nous aurions un Président de la République et un Premier ministre qui découvriraient ce que tous les parlementaires savaient

en était. Monsieur le Premier ministre, vous étiez pourtant, comme M. le ministre de l'économie et des finances, membre du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Or notre excellent collègue Gilles Carrez, alors président de la commission des finances, avait, à l'automne dernier, alerté sur l'insincérité du budget 2017. Je ne doute pas qu'à l'époque vous l'écoutiez avec attention. Ici même, au Sénat, notre rapporteur général, Albéric de Montgolfier, avait fait de même et la majorité sénatoriale avait repoussé ce budget, refusant de l'examiner en séance-mais pas en commission

Je pense que nos concitoyens l'ont bien compris : la hausse de la CSG et du prix du tabac, c'est pour tout de suite ; les baisses d'impôts et de charges, ce sera pour plus tard. La première décision de tout gouvernement constatant une telle situation aurait dû être de présenter un collectif budgétaire, dans l'esprit de la LOLF. Vous vous y refusez. trente-deuxième loi de moralisation de la vie publique ... Vous allez donc tenter de contenir le déficit 2017 à coup de nouveaux gels ou de surgels de crédits-Didier Migaud nous a dit lors de son audition que le congélateur était plein et qu'il fallait en finir avec ces pratiques.

Pour autant, on comprend bien que, pour vous, cette technique a l'immense avantage d'éviter un débat devant le Parlement, et donc devant les Français. Je pense que vous faites là une erreur. Autre sujet de préoccupation, particulièrement ici au Sénat : vos annonces concernant les collectivités locales. On avait cru comprendre, d'après ce qu'avait dit Emmanuel Macron au cours de la campagne, qu'il n'y aurait plus de baisses des dotations de l'État, le Président souhaitant en contrepartie une baisse de nos dépenses de 10 milliards

La suppression annoncée de la taxe d'habitation pour 80 % des Français pose un vrai problème, peut-être même constitutionnel. La taxe d'habitation est, avec la taxe foncière, la dernière ressource propre des communes. Couper ce lien fiscal entre le citoyen et sa commune, c'est d'un côté amoindrir la responsabilité des élus, leur ôter tout pouvoir de taux, et de l'autre entamer un peu plus l'autonomie financière de ce qui reste, n'en déplaise à certains, la cellule de base de notre démocratie. Chacun reconnaît que les modes de calcul de la taxe d'habitation comme de la taxe foncière sont obsolètes et profondément inéquitables. Voilà pourquoi il est urgent de mener à bien la réforme des valeurs locatives : si le système est injuste, vous ne pouvez pas le faire perdurer pour 20 % des contribuables, d'autant que la taxe foncière est assise sur les mêmes bases. Tout à fait ! Il nous faut donc cette réforme des valeurs locatives

car il n'est plus possible de toucher à l'une sans toucher aux autres. Monsieur le Premier ministre, après la baisse de 11 milliards d'euros des dotations que nous avons subie depuis 2014, les élus locaux sont encore prêts à des efforts mesurés, mais ils ne veulent pas se trouver sous perfusion de dotations d'État, dont on sait qu'elles finissent toujours par être la variable d'ajustement de tout le reste, pas plus qu'ils ne veulent d'un nouveau big-bang institutionnel. Les élections présidentielles et législatives ont une nouvelle fois mis en évidence la double fracture, territoriale et sociale, qui traverse notre pays.

Il y a bien une France qui ne va pas trop mal, qui profite des opportunités de la mondialisation : celle des cadres, des CSP+, des centres-villes, des métropoles, des régions qui voient leur population augmenter. Puis il y a une France rurale, celle des agriculteurs qui peinent à se payer un salaire, celle des territoires en voie de désertification, mais aussi la France des banlieues en difficulté, celle des ouvriers qui voient la désindustrialisation se poursuivre, La France de tous ceux qui se sentent les perdants de la mondialisation. L'écart entre ces deux France n'a jamais été aussi grand et continue de se creuser. À ceux qui ne voient, dans le résultat de la présidentielle et, peut-être plus encore, dans celui des législatives, que le triomphe d'une nouvelle génération d'élus sur l'ancienne, je dis : prenez garde Jamais autant de Français-ils ont été 40 % au premier tour de la présidentielle -ne s'étaient tournés vers des candidats proposant de renverser la table. Jamais autant de Français ne s'étaient abstenus pour des élections législatives. C'est autant à eux-et peut-être plus à eux qu'aux autres -que vous devez répondre, monsieur le Premier ministre. Votre responsabilité est immense et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Quant à nous, comme la majorité sénatoriale l'a toujours fait, nous assumerons nos responsabilités, dans le calme et la sérénité. Si vos décisions nous semblent aller dans le bon sens, nous vous accompagnerons si c'est l'inverse, bien évidemment nous nous y opposerons. C'est aussi cela une démocratie : une majorité et une opposition.

Vous avez la parole, vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'après trois discours nous ne sommes toujours pas convaincus que la politique que vous nous proposez va résoudre les problèmes qui touchent nos compatriotes- insécurité, immigration subie et chômage de masse, pour ne prendre que les trois plus importants -et qu'elle risque également d'aggraver la dissolution progressive de notre pays et de notre civilisation dans un magma mondialisé. Après un discours présidentiel totalement déconnecté de la réalité vécue par l'immense majorité des Français, nous avons celui d'un gestionnaire, comme si l'action politique se limitait à une simple vision comptable Il faut dire que, dans ce domaine, la situation n'est pas brillante, après les deux derniers quinquennats, la dette de notre pays ayant bondi de 600 milliards d'euros sous M. Sarkozy, alors soutenu par votre famille politique d'origine, monsieur le Premier ministre, et de 340 milliards d'euros sous M. Hollande, dont l'actuel Président de la République a été le conseiller puis le ministre. Après une décennie d'austérité imposée par l'Union européenne, vous nous proposez la même chose ! Il faut dire que, n'ayant pas récupéré une once de souveraineté, vos leviers d'action sont bien limités. Ainsi, votre objectif est non pas de faire baisser le chômage, qui touche plusieurs millions de nos compatriotes, mais d'abord de respecter la règle maastrichtienne des 3 % pour obéir aux commissaires bruxellois. Les caisses sont vides ? Qu'à cela ne tienne, vous augmentez les impôts : CSG, cigarettes, diesel ! Certes, vous patinez certaines hausses de bons sentiments, mais en réalité le but est juste de faire rentrer de l'argent sans avoir à changer de modèle. Et ce sont encore les classes moyennes qui vont subir de plein fouet cette austérité. Quant aux différentes promesses pour le pouvoir d'achat, aux baisses de charges pour les entreprises, notamment les TPE, à la défiscalisation des heures supplémentaires, on verra plus tard ! La vérité est que vous devez attendre que la Commission européenne donne son feu vert. En revanche, certains lobbys se frottent les mains, l'industrie pharmaceutique, par exemple, après que vous avez annoncé l'augmentation considérable du nombre de vaccins obligatoires. Au fait, vous êtes-vous demandé pourquoi des maladies disparues de notre sol depuis longtemps refaisaient surface ? Il faut avoir le courage de dire que l'immigration massive est la meilleure piste de réponse Même au niveau européen, vous soumettez les Français à ces lobbys, si j'en crois la position récente de la France sur les perturbateurs endocriniens, première couleuvre pour le ministre d'État Hulot D'ailleurs, permettez-moi de relever que l'écologie a été bien vite balayée dans votre discours. Il faut dire que le combat écologique, qui doit être intégral, c'est-à-dire, environnemental, économique et social, se marie mal avec le modèle de développement que vous vous évertuez à défendre. Pourtant, des mesures simples pourraient être prises la mise en place du patriotisme économique pour les produits agricoles, le refus des traités de libre-échange ou encore la création d'une véritable filière d'énergies renouvelables, grâce à la priorité donnée aux entreprises nationales du secteur. Autres grands absents de votre discours, et c'est extrêmement inquiétant : la sécurité et l'immigration. À part le fait de faire entrer un état d'exception, l'état d'urgence, dans le droit commun : rien ! Alors que, pour renforcer la sécurité de nos compatriotes, il y a tant de mesures à mettre en oeuvre, notre droit vous donnant déjà pas mal de possibilités-par exemple appliquer l'article 411-4 du code pénal -, ou de mesures à prendre : contrôles systématiques aux frontières, fermeture de la centaine de mosquées radicales, expulsion des étrangers fichés Sur l'immigration, et l'enchaînement n'est évidemment pas fortuit, n'en déplaise aux ténors du politiquement correct : rien non plus ! Enfin, comme tant d'autres avant vous, vous promettez une réforme du droit d'asile. J'étais encore enfant que votre mentor, M. Juppé, disait déjà la même chose.

et lutter beaucoup plus efficacement contre les passeurs, surtout quand ceux-ci sont déguisés en ONG ! Pas un mot non plus sur le communautarisme qui gangrène nos quartiers et qui fait que certains de nos compatriotes ne se sentent plus chez eux, une culture-voire une loi -étrangère ayant remplacé la civilisation française. Concrètement, que faites-vous pour que dans les rues de notre capitale, une femme puisse se promener sans avoir à-je cite -« tenir son sac et baisser les yeux » ? Avant de conclure, un mot sur une annonce discrète, mais symbolique. Nous avons bien senti ici, dans cette chambre représentant les collectivités, que vous comptiez vous attaquer aux communes, symbole de notre pays, en les diluant davantage dans des intercommunalités, d'ailleurs transférer de nouvelles compétences, et en enlevant encore aux maires certaines prérogatives. Les Français sont attachés à leur commune et à l'image du maire, serviteur public de proximité. Soyez sûr que toute tentative de vous attaquer à ces symboles sera fermement combattue. Vous marchez, mais vous ne savez pas vers où. La marche vous suffit. Mais le flou de votre discours, dans la lignée du flou de la campagne, risque de ne pas résister longtemps au monde réel. Soyez sûr que nous serons là pour vous rappeler la réalité et pour combattre toute mesure qui n'aura pas pour objectif de protéger nos concitoyens, de défendre les plus fragiles d'entre eux et de réarmer économiquement et moralement la nation française.

parce qu'il n'y aura pas d'état de grâce, parce que le Gouvernement doit réussir, monsieur le Premier ministre, vous pouvez être assuré du soutien que vous apportera, aujourd'hui et demain, durablement, le nouveau groupe sénatorial La République en marche. me permettrez de saluer l'initiative du Président de la République pour son adresse solennelle dès le début de la législature à toute la représentation nationale et, à travers nous, à tous nos concitoyens de l'Hexagone et d'outre-mer-les outre-mer sont particulièrement bien représentés au sein de notre groupe, ce dont je me réjouis. Le soutien actif des sénateurs de La République en marche répond à trois motifs essentiels. le Premier ministre, vous avez parfaitement dissipé l'ambiguïté que certains voyaient ou feignaient de voir dans la succession rapprochée de deux interventions capitales, celle du Président de la République lundi et la vôtre hier. On avait même parlé d'effacement du Premier ministre au profit du Président. Il y avait dans cette critique un double paradoxe. Elle était émise par ceux qui se réclament volontiers du général de Gaulle des institutions qu'il a données à notre pays. Or les deux têtes de l'exécutif ont donné une lecture parfaite de la Constitution, de sa lettre et plus encore de son esprit. Il appartient au Président de fixer le cap, de proposer un horizon ; et il est de la compétence du Premier ministre de définir la politique à mettre en oeuvre par le Gouvernement pour assumer cette ambition. C'est le partage des tâches auquel les Français sont légitimement attachés, l'appliquez très exactement. L'autre partie du paradoxe, nouveau reproche par anticipation adressé au Président, repose sur une accusation à l'égard d'un discours-programme très détaillé et concret qui entrerait dans votre compétence et non dans la sienne. Sans trop de souci de cohérence, les mêmes ont adressé au Président, dès lundi soir, un reproche systématiquement inverse : il nous aurait livré une allocution trop vague, trop générale, trop « philosophique trop générale, trop « philosophique »-j'ai découvert, à cette occasion, que l'adjectif « philosophique » serait devenu péjoratif ... Le Président Macron nous a en effet livré sa vision de la politique, une vision très élevée, exigeante, qui constitue bien une véritable philosophie du pouvoir. Je répondrai à ces détracteurs systématiques que, philosophie pour philosophie, ils auraient dû relire, comme le Président l'a fait, Héraclite d'Éphèse, qui disait : « On n'entre jamais deux fois dans le même fleuve. » Eh bien, mes chers collègues, on n'entend jamais deux fois le même discours.

vous avez montré le cap, exprimé la vérité en vue d'obtenir des résultats concrets et rapides dans les domaines de la sécurité, de l'économie, de la santé, de l'éducation, du logement, de la transition écologique ou encore de l'aide aux plus démunis. c'est un fait politique nouveau : le Gouvernement tiendra les engagements qu'il a pris. Nous vous accompagnerons, même quand il faudra rechercher l'adhésion du pays dans la réalisation du programme, courageux et indispensable, de réduction de la dépense publique et du déficit que vous avez annoncé. En troisième lieu, nous avons apprécié dans vos propos le rappel des grands principes de la méritocratie républicaine à propos de l'école, de l'université, de la formation professionnelle, de l'aide à la création d'entreprise. Vous préférez le principe de justice à celui, théorique, de l'égalité, car ce mot est source de malentendu. Nous voulons l'égalité des droits et des chances quand d'autres rêvent de l'égalité des situations, qui est toujours hélas ! synonyme de nivellement par le bas. Nous sommes, au sens propre, d'une autre école. Aidés par les meilleurs élèves, nos maîtres tendaient la main aux plus faibles, aux moins favorisés pour les faire aller plus vite et plus haut. Telle est notre vision de l'avenir de ce pays. Nous voulons libérer toutes les initiatives et les projets de ceux, innombrables, dont les entreprises illustrent le génie particulier de ce pays. Et dans le même temps, la responsabilité des pouvoirs publics, de l'État, mais aussi des collectivités territoriales et de l'Europe sera de garantir aux autres l'égalité des chances. Nous voulons une société qui libère et qui protège. Nous venons de vivre deux de ces grandes journées qui honorent une nation lorsqu'elle décide de ressembler au meilleur d'elle-même. Il est des révolutions-et ce sont les plus admirables -qui s'opèrent sans violence, simplement parce que la volonté des hommes libres s'oppose à la fatalité. D'autres avaient cru entendre un simple slogan, mais nous le voyons aujourd'hui : notre République est véritablement en marche. L'exigence de nos concitoyens nous oblige, Gouvernement et Parlement, au volontarisme comme à la réussite. Nous, députés et sénateurs de La République en marche, devons être à la hauteur de ce moment. Il est l'heure, mes chers collègues, de transformer notre République, de la moderniser, de la refonder, de lui donner un horizon, de bâtir une France nouvelle. Les Français doivent retrouver fierté et confiance. Le Président a défini un projet ambitieux pour notre nation. Nous sommes prêts et déterminés. Déterminés à agir Déterminés à agir pour le vivre ensemble et l'intégration, la cohésion nationale. L'éducation et la culture sont au coeur de notre projet de société tout comme la laïcité, qui ne saurait plus longtemps être galvaudée pour être tantôt bouc émissaire, tantôt stigmatisation. La laïcité est le ciment de notre démocratie et la protéger est notre dessein. Déterminés à lutter contre le chômage de masse, à former les plus éloignés de l'emploi, à moderniser et à simplifier le droit, à réformer l'assurance chômage pour en faire un droit universel, à améliorer le pouvoir d'achat de chacun. Déterminés à moderniser notre économie grâce à une stratégie d'investissement ambitieuse dans tous les territoires urbains, certes, mais également ruraux. J'y tiens tout particulièrement. Les territoires Les territoires ultramarins ne devront pas être oubliés-vous les avez d'ailleurs cités, monsieur le Premier ministre. Pour ce faire, la France devra proposer un projet d'émancipation réelle des outre-mer, tout en reconnaissant leur légitimité à avoir des règles adaptées à leurs réalités locales, notamment un taux de chômage nettement supérieur à la moyenne nationale, en particulier chez les jeunes, et un coût de la vie plus élevé. Ils Ils veulent l'équité pour pouvoir réussir là où ils sont dans la République. Déterminés à mettre en oeuvre un modèle de croissance réconciliant transition écologique, industrie du futur et agriculture de demain. Déterminés à garantir la sécurité de nos concitoyens, à restaurer partout l'autorité de l'État, à affronter le terrorisme. Déterminés à repenser notre démocratie, à développer la participation citoyenne, à garantir la respectabilité de nos élus. Déterminés à défendre les intérêts de la France et à relancer le projet européen, celui d'une Europe qui protège et qui investit. Ces chantiers sont nombreux pour bâtir cette France que nous appelons de nos voeux. Mais nous sommes des millions à vouloir la construire, pour donner des perspectives aux enfants de la France, la France des Lumières et des droits de l'homme.

Nous avons beau tendre l'oreille, ce n'est pas le souffle du renouveau que nous entendons, mais des refrains usés, et la nouvelle orchestration n'y change rien. Le macronisme était, paraît-il, une révolution. Versailles a remis les pendules à l'heure.

d'abord fallu envoyer un signal clair de rupture avec la dérive présidentialiste de notre régime : cet anachronisme qui consiste, au XXI siècle, à concentrer toujours plus de pouvoirs dans les mains du seul Président de la République. Il aurait fallu dire aux Français : « Nous allons vous rendre du pouvoir, instaurer de nouveaux droits d'intervention des citoyens dans toutes les décisions et de nouveaux droits des salariés dans les entreprises, pour que ce ne soient plus les seuls intérêts de la finance qui décident. » Voilà qui aurait été une entrée en matière révolutionnaire ! Il aurait fallu adresser un signal de confiance au Parlement, et non une convocation à Versailles, un discours monarchique où le Président parle et, tel un monarque, se retire, non sans avoir signifié aux parlementaires qu'ils sont trop nombreux et laissé entendre que le Conseil économique, social et environnemental

Nous avons combattu ici même un monstre législatif de 400 articles, ... Eh oui ! ... tous écrits sous la dictée des intérêts patronaux, la fameuse loi Macron adoptée par 49.3, ... Exact ! ... celle qui, aujourd'hui, oblige à travailler le dimanche, qui autorise la privatisation de nos aéroports régionaux, qui facilite les licenciements, qui a affaibli l'inspection du travail, et j'en passe. Oui, voilà des lois dont les Français ne voulaient pas. Monsieur le Premier ministre, comptez donc sur nous pour résister à l'inflation législative produite par les lobbys des grands intérêts capitalistes et pour multiplier les propositions qui redonneront du pouvoir aux citoyens. Mais ne comptez pas sur nous pour faire allégeance à une dérive autoritaire de nos institutions. Vous voulez d'ailleurs, pour commencer, casser le code du travail en nous privant du débat parlementaire qu'appelle un tel chantier. Nous voterons contre l'habilitation à procéder par ordonnances. Nous ne nous dessaisirons pas de notre pouvoir légitime de légiférer en la matière et nous ferons tout pour révéler aux Français le contenu de ces projets. L'été, symbole des congés payés gagnés de haute lutte, n'est pas fait pour casser le code du travail dans le dos de ceux qui suent au labeur toute l'année et qui prennent alors un repos légitime. Très bien Pour rendre au pays l'espoir auquel il aspire, pour inventer un nouvel avenir social, productif et écologique, il ne faut pas, comme vous l'avez dit hier, désintoxiquer le pays de la dépense publique. Sous le quinquennat précédent, l'investissement public a chuté de 25 %, et pour quel résultat ? En réalité, il faut désintoxiquer le pays de la finance, de la prédation des richesses communes par les exigences d'une rentabilité financière à courte vue. Vous ne dites rien de l'évasion fiscale, qui coûte 80 milliards d'euros par an au pays, rien de la résolution votée sur notre initiative par l'Assemblée nationale pour une COP fiscale mondiale, rien de l'explosion des 500 premières fortunes professionnelles françaises, rien du rôle défaillant des banques et de leurs critères de crédit. Et vous parlez de moraliser la vie publique ! Mais l'indécence de l'argent crève les yeux, et c'est à elle qu'il faut s'attaquer. Bien au contraire, vous proposez d'en rajouter, toujours prétendument au nom de l'emploi : allégement de l'impôt de solidarité sur la fortune, baisse de l'impôt sur les sociétés, transformation du CICE en baisse de cotisations patronales pérennes.

de « ceux qui sont installés », de ceux qui ne devraient pas se résoudre à être des assistés. Mais savez-vous vraiment de qui vous parlez ? Au total, neuf millions de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté à cause du chômage et de la précarité engendrée par le modèle économique actuel, que vous défendez. Plutôt que de casser le code du travail, nous vous demandons d'inscrire à l'ordre du jour du Parlement notre proposition de loi pour une sécurité de l'emploi et de la formation. nous vous demandons la convocation de deux grandes conférences sociales relatives, l'une, au relèvement des salaires et des qualifications, l'autre, à la lutte contre l'exclusion et la grande pauvreté, demandées par toutes les associations qui se consacrent à ces questions, pour définir des plans d'action cohérents et pluriannuels. Oui, dans ce pays, on ne doit plus travailler pour un salaire de misère, on ne doit plus être expulsé de son logement parce qu'on ne parvient plus à le payer. Dans votre discours d'hier, vous avez fustigé les aides au logement. Mais le pays manque cruellement d'aides à la construction de logements sociaux et accessibles à tous. Il manque cruellement de fonds publics dédiés à la rénovation thermique de l'habitat.

La France rend aujourd'hui hommage à Simone Veil. Soyons à la hauteur de l'audace qui fut la sienne et, quarante ans après la loi qui porte son nom, franchissons une nouvelle étape. Nous proposons qu'à la faveur de la réforme constitutionnelle qui s'annonce le droit à l'interruption volontaire de grossesse soit désormais inscrit dans notre Constitution. La cause des services publics est un autre pilier de la lutte pour l'égalité. Vous n'annoncez aucun nouveau moyen pour l'école. En fait, vous encouragez un pragmatisme et une autonomie des établissements qui masquent la mise en cause de l'unicité de notre système éducatif. Ce faisant, vous renoncez à la lutte contre les inégalités. En matière de santé, derrière vos annonces relatives aux vaccinations ou la promesse de meilleurs remboursements forfaitaires pour les lunettes ou les aides auditives,

Ce qui aurait été réellement innovant, en rupture véritable avec les quarante dernières années, c'est un grand plan d'investissement pour les services publics, pour le développement industriel et pour la transition écologique. Vous annoncez un plan de 50 milliards d'euros, une somme qui sonne rond, mais qui est bien dérisoire au regard des enjeux

Refusons le fossé qui se creuse, nous dites-vous. Soit, mais comment agir sans une ambition d'égalité sur tout le territoire, sans un moratoire immédiat des réductions de dotations et des fermetures de services publics pour que plus un seul habitant de notre pays, qu'il vive dans un quartier populaire, en zone rurale ou dans la périphérie des villes, ne se sente abandonné, délaissé, méprisé, tel un citoyen de seconde zone Vous annoncez une conférence des territoires : parfait. Mais pour quoi faire ? Pour réduire à deux, sous les régions, les niveaux de collectivités, avez-vous dit. Traduisons : cela signifie ou la mort des départements, ou le regroupement massif de communes qui seraient d'ailleurs privées de leurs compétences d'urbanisme.

Conscient vous-même de l'impasse dans laquelle vous conduisez la plupart des communes, vous commencez à tergiverser quant à la suppression de la taxe d'habitation, ce pour une raison simple : vous ne savez pas comment compenser cette perte de revenus mortelle pour les communes.

Il est temps d'entrer dans un nouvel âge, de donner aux collectivités d'outre-mer les moyens de maîtriser leur avenir, avec plus de responsabilités et plus de compétences, et avec un fonds de développement pour bâtir un projet durable et cohérent en matière sociale et écologique. Ne manquons pas ce rendez-vous avec l'histoire. Enfin, être à la hauteur de l'époque serait faire de la France une grande messagère de la paix et de la solidarité dans le monde. Au lieu de cela, vous nous annoncez l'inscription des dispositions de l'état d'urgence dans notre loi commune et une augmentation à 2 % du PIB des dépenses militaires. Par ces mesures, le N'est-ce pas là, d'ailleurs, la véritable raison de l'invitation de Donald Trump, le 14 juillet prochain, à Paris ? J'imagine que ce n'est ni sa volonté de fêter avec nous la prise de la Bastille ... Si, si ! ... ni son action révolutionnaire contre le réchauffement climatique qui lui vaut cette invitation. Monsieur Monsieur le Premier ministre, vous avez salué hier le courage tranquille des Français. C'est un de nos rares points d'accord. Comptez sur nous pour donner aux Français le courage de rêver et de continuer à agir pour un monde meilleur. Hier, vous avez

connaît à la fois la dureté de l'histoire et la dureté des transformations économiques. Cette ville, c'est la mienne, j'en suis fier, et je vous remercie de m'avoir permis de le dire devant le

rapport de la Cour des comptes ne m'a pas mis en colère. Plus exactement, il ne m'a pas donné envie de rechercher des coupables, et je ne suis pas sûr qu'il nous faille rechercher des coupables. En tout cas, tel n'est pas le terrain sur lequel je me place.

Nous ne faisons pas de collectif budgétaire. Nous indiquons que nous allons tenir, dès 2017, l'objectif de 3 %. Pourquoi 3 % ? Parce que c'est un engagement qui a été souscrit par la France- mais par la France. Cet engagement a été pris depuis longtemps et, depuis longtemps, il n'est pas tenu, pour des raisons qui peuvent s'expliquer et qui peuvent même se justifier à certains égards. Mais reconnaissons là aussi, tranquillement- entre nous, si j'ose dire que tous les pays confrontés aux mêmes difficultés que nous ont fait les efforts nécessaires pour revenir sous le seuil qu'ils avaient librement accepté de respecter vis-à-vis de leurs partenaires. Nous sommes les derniers,

et charge les générations à venir, nos enfants et nos petits-enfants, de la responsabilité de rembourser les dettes, c'est-à-dire ce que nous ne voulons pas payer pour nous-mêmes.

les impôts et de contenir le déficit en réduisant les dépenses. C'est un objectif ambitieux, mesdames, messieurs les sénateurs, mais nous allons l'atteindre

En 2018, nous augmenterons la CSG en contrepartie d'une diminution des charges ainsi que des cotisations salariales et sociales. C'est là un choix politique, qui ne devrait étonner personne : il a été présenté pendant la campagne électorale,

Tous ceux qui connaissent les finances municipales savent combien l'impossibilité de moduler, en fonction des quartiers, un certain nombre de taux tend à accroître dans la durée